J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.

Aux termes de la loi relative à la bioéthique du 7 juillet 2011, l'accès aux techniques de l'assistance médicale à la procréation (AMP) est réservé aux couples homme-femme, vivants, en âge de procréer, le caractère pathologique de l'infertilité étant médicalement diagnostiqué. Il est donc nécessaire d'identifier clairement les causes pathologiques qui motivent le recours à l'AMP, car elles permettront d'emprunter de nouvelles pistes dans la recherche sur l'infertilité. De plus, l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules risque de se traduire par un accès beaucoup plus difficile pour les couples hétérosexuels, dans un contexte de levée de l'anonymat, qui entraînera un tarissement des dons de sperme, comme cela a pu être vérifié au Danemark. Il importe donc de s'assurer que les couples hétérosexuels ne seront pas victimes d'une discrimination.

une approche méthodologique qui nous semble présenter de nombreux avantages par rapport à tout autre type d'études qui pourrait être proposé. Je pense notamment au suivi anonyme des personnes tout au long du parcours de soins, à la représentativité

le remboursement partiel de cet acte est justifié par le fait qu'il s'agirait d'une technique de médecine préventive pour la prévention de l'infertilité, ce qui n'est pas sans poser de question. Ce qui m'interroge n'est pas tant le remboursement

agissons en conséquence et mettons nos gamètes à l'abri, pour y revenir ultérieurement sans qu'ils aient été altérés par l'environnement dans lequel nous En outre, j'ai des doutes sur les motivations réelles des personnes qui auront recours à cette méthode : se préoccuperont-elles vraiment d'une infertilité probable ? Je ne le pense pas ! Elles agiront souvent sous la pression

à ces problématiques, je m'interroge sur la fausse bonne idée que pourrait représenter cette mesure d'autoconservation de gamètes. Dans quelle logique s'inscrit-elle au regard de l'émancipation des femmes ? Dans quelle mesure pallie-t-elle pallie-t-elle nos inactions en matière de politique familiale et environnementale ? Et je ne parle pas de la mesure visant à ouvrir aux établissements privés à but lucratif la possibilité de conserver les gamètes en question

Par ailleurs, le nombre de donneurs devrait augmenter du fait de l'autorisation de l'autoconservation. Je suis donc favorable à ce que les établissements privés à but lucratif soient autorisés à pratiquer des activités de conservation des gamètes, en complément de l'offre publique et privée sans but lucratif.

La durée des études, l'inscription dans la vie active, la recherche d'une stabilité financière, la construction d'une vie amoureuse et d'un projet parental conduisent les femmes à avoir des enfants de plus en plus tard.

se réaliser, il s'agit de permettre aux femmes et aux hommes de conserver leurs gamètes, afin qu'ils puissent différer leurs projets d'enfants. Certaines femmes pourraient ainsi s'affranchir d'un choix que leur imposerait notre société

Certains médecins, en France, prescrivent illégalement les traitements et les examens, en vue d'une congélation qui aura lieu à l'étranger. Certains vont même jusqu'à pratiquer le prélèvement et la congélation pour les patientes qui n'entrent pas dans le cadre autorisé par la loi. Aux termes l'article 2, il ne s'agit pas d'encourager la congélation massive d'ovocytes. Nous le savons, c'est un acte lourd, qui nécessite de stimuler les ovaires avec un traitement hormonal, par le biais d'injections quotidiennes pendant une douzaine de jours. Cela implique des échographies de contrôle, des prises de sang tous les deux jours et, enfin, la ponction d'ovocytes sous anesthésie locale ou générale. Personne ne prend ce genre de décision à la légère

que de prendre en charge des décisions de pure convenance personnelle ou, pire encore, de faciliter les besoins de l'entreprise ? En outre, est-ce la vocation de

de porter un enfant quand on le souhaite. Quand on offre, par la science, des possibilités de différer une grossesse, on prend une lourde responsabilité d'ordre sociétal. Cette

n'est pas un handicap dans le milieu du travail ? Le fait que les femmes portent les enfants, c'est l'avenir de la société, pas seulement celui du régime de retraite par répartition. Pourtant, la grossesse n'est pas considérée

Nous sommes effectivement aujourd'hui confrontés à un recul de l'âge à la naissance du premier enfant, qui est la conséquence d'un mouvement d'ampleur et qui ne devrait pas s'inverser dans les années à venir, parce qu'il résulte de changements considérables qui sont survenus dans les comportements au cours des dernières années.

dans la mesure où les propres ovocytes de la femme conservés antérieurement seront utilisés, d'autre part, d'augmenter les gamètes disponibles pour le don dans l'hypothèse où, n'en ayant pas eu besoin, les femmes et les hommes concernés les donneraient finalement pour qu'ils bénéficient à d'autres femmes et à d'autres hommes. S'agissant de la question de la fertilité, qui a été évoquée par un certain nombre d'entre vous, l'autoconservation est bien une mesure supplémentaire en faveur de la fertilité. Néanmoins, elle ne garantit pas une naissance et il sera avant tout important de mieux informer la population sur les enjeux de la fertilité. Le Gouvernement a eu l'occasion de s'engager à cet égard devant l'Assemblée nationale. Tel était également l'objet des débats que vous avez eus

offerte aux femmes et la nécessité de prévoir un certain nombre de garde-fous pour qu'il ne soit pas porté atteinte à d'autres principes fondamentaux de notre droit et de notre société. Pour toutes ces raisons, et parce que ce principe-là ne contrevient à aucun principe bioéthique, nous estimons que cet article 2 a évidemment toute sa place au sein de ce projet de loi.

Je ne crois pas à la vision rousseauiste de la société ; je ne crois pas à la bonté d'âme au-dessus de tout ; je crois que, malheureusement, et on le voit tous les jours et à tous les niveaux,

La vérité, c'est que nous vivons dans des sociétés, en des temps où, malheureusement, le commerce, la marchandisation, la pression sont réguliers. Et je dis tout de suite

Donc, en la matière, je n'ai pas beaucoup de leçons à recevoir. Quel modèle de société veut-on ? J'ai voté l'article 1 parce que j'avais le sentiment qu'il n'était pas juste que des gens aient le droit à la PMA et d'autres pas.

Moi, j'aime la société française telle qu'elle est. Elle peut évoluer, elle doit évoluer, mais laissons-la humaine.

Je voterai également ces amendements de suppression parce que, comme le disait M. Karoutchi, je pense que, malheureusement, nous ne sommes pas dans un monde parfait et que la pression sociale des entreprises notamment pourrait s'exercer en faveur de cette autoconservation des gamètes. On le sait, le monde de l'entreprise est un monde dur, c'est un monde de pouvoir, c'est parfois, et l'actualité le démontre, le lieu du harcèlement, de la pression sur les individus. Il existe bien du mal-être au travail, et l'on ne peut pas le négliger.

qui ont besoin de stabilité, qui ont besoin de performances, qui ont besoin d'un engagement total de leurs salariés, surtout quand ils occupent des postes à haute responsabilité. En quelque sorte, elles ont besoin de passer un contrat de confiance

mais il n'est ni tout noir ni tout blanc. Ce qu'a cherché à faire la commission spéciale, c'est tenir compte des nuances de notre société, de l'évolution sociétale qui est en marche. Mais on peut aussi changer

de vote. Élisabeth Doineau a bien rappelé que le texte dont nous discutons prohibe tout financement

la bioéthique, c'est qu'il faut à la fois associer des techniques médicales et scientifiques nouvelles avec des valeurs qui, parfois, sont aussi orthogonales entre elles.

prendre ou non un moyen de contraception, choisir ce moyen- nous nous battons contre l'injonction à la contraception unique qui pèse sur les femmes. Tout ce que ce texte propose, c'est de laisser aux femmes le choix.

que les droits des femmes ont progressé, que ce soient leurs droits civils, civiques ou procréatifs, chaque fois on nous a annoncé une catastrophe pour la civilisation, chaque fois cela a été la même histoire. Quand les femmes

d'une autoconservation ovocytaire apparaîtrait comme un espace dans lequel la liberté des femmes pourrait s'exercer sans qu'elles compromettent leur maternité future

à l'autoconservation des ovocytes ! Il s'agit simplement d'ouvrir un droit en créant un dispositif qui est très encadré par la commission spéciale.

il ne faut jamais faire à une opinion l'honneur de l'intolérance. Je vous

Je suis, moi, un humble médecin ; je fais de l'imagerie de la femme, et mon avis a changé depuis que je suis près des femmes qui désirent procréer. Ce qui me gêne, c'est de légiférer sur ce que la femme a le droit de faire de son corps.

une telle chance d'accomplissement pour soi-même, dans le fait de pouvoir être père ou mère, que préserver les chances de chacun de l'être un jour est un objectif noble.

Et j'ai peur que l'on crée, à travers une forme d'épargne d'ovocytes, une fausse sécurité. J'ai peur qu'on donne l'illusion qu'est possible une sorte d'assurance grossesse. Il n'en est rien Car la difficulté de la grossesse, à mesure que l'on avance en âge, ne tient pas uniquement au nombre et à la qualité des ovocytes dont on est porteuse. Il ne faut pas répandre l'illusion selon laquelle, parce qu'on aura mis de côté des ovocytes, on pourra avoir un enfant. Cette illusion est dangereuse.

les amendements de suppression. Je dois dire que je ne m'y suis pas décidé d'entrée de jeu : je trouve la question vraiment difficile.

Il est arrivé que la communauté scientifique se mette d'accord sur des limites- Bruno Retailleau parlait hier d'interroger les limites avant d'en fixer.

les couples se forment bien plus tard, et la durée de vie est telle que les femmes ne réalisent pas forcément aujourd'hui que des problèmes de fertilité pourraient se poser.

cette autoconservation pour d'autres raisons que des raisons médicales, c'est parce qu'elle a constaté l'évolution de la société, qui a été décrite par les uns et par les autres

autant de questions qui sont au coeur des réflexions et des travaux que nous menons en ce moment, et dont vous avez connaissance, autour de cette période cruciale pour l'enfant que ce sont les mille premiers jours

aux propos tenus dans l'assemblée, en l'occurrence aux miens, que la liberté de parole est un des privilèges individuels fondamentaux des droits des parlementaires. Sans la liberté de parole des parlementaires, il n'y a pas de démocratie parlementaire, il n'y a pas de liberté de conscience, il n'y a pas de liberté d'opinion et il n'y a pas de liberté d'expression ! Comme chacun d'entre vous dans cette assemblée, je suis en droit d'exprimer mes opinions,

du temps où les femmes étaient considérées comme des incapables majeures, de l'assignation à la procréation, de l'interdiction de la contraception et de l'avortement, de l'interdiction d'exercer leurs droits civiques, tous nos droits ont été conquis progressivement.

en 2011. Supprimer l'exigence que les donneurs aient déjà procréé n'a rien d'anodin et donner ses ovocytes sans avoir procréé présente certains inconvénients. Tout d'abord, lorsque le donneur n'a pas procréé, il ne peut réaliser la portée de son geste. C'est le fait d'avoir déjà procréé qui permet de consentir en connaissance de cause. Les conditions de l'expression d'un consentement libre et éclairé ne paraissent donc pas réunies. Ensuite, accepter le don de gamètes de personnes n'ayant pas procréé risque de susciter chez le donneur des conséquences psychologiques graves allant de la préoccupation jusqu'au fantasme nourri à propos des enfants issus du don, notamment

? Sans vouloir raviver le débat que nous venons d'avoir, si nous réintroduisons la condition pour le donneur d'avoir procréé,

Il me semble, mais cela ne vous étonnera pas, puisque nous parlons de ce sujet depuis maintenant plusieurs heures, que chaque être humain- il ne s'agit pas que des femmes -doit être libre de disposer de son corps.

depuis. Nous partageons l'idée que le don de gamètes engage chacun personnellement. Que le donneur tienne informé son conjoint ou sa conjointe, dans le cadre d'un PACS, d'un mariage ou d'un concubinage, c'est très bien, mais cela relève de la sphère privée et non de la loi. On a le droit, même si on est en couple, de prendre des décisions individuelles. Je vous souhaite d'ailleurs qu'il en soit ainsi dans vos couples respectifs ! C'est vraiment une remarque inutile ! Par ailleurs, il est nécessaire d'adapter le don de gamètes aux évolutions de la société et de le sécuriser en permettant au seul donneur de gamètes de révoquer son consentement. Nous aurons l'occasion d'y revenir l'occasion d'y revenir à l'article 3, avec un amendement visant à supprimer le recueil du consentement de l'autre membre du couple dans le cadre de l'accès à l'identité

explication de vote. Je ne comprends pas le postulat qui a été posé dans plusieurs interventions et qui consiste à dire que le don a une incidence sur la vie du couple. Quelle incidence le don a-t-il sur la vie du couple ?

Dans la mesure où la commission spéciale a accepté de lever l'anonymat des donneurs de gamètes, son avis est nécessairement défavorable.

à une pénurie de gamètes et, donc, à la tentation de la commercialisation.

du Gouvernement, qui prévoit de fixer par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, les conditions d'âge pour autoconserver ses gamètes. Il est indispensable d'enserrer la réforme dans des conditions strictes d'accès en termes d'âge pour ne pas

des gamètes prélevés ou recueillis, un âge supérieur doit également être fixé. À défaut, ce serait une perte de chance pour les personnes concernées. Si des limites chiffrées n'étaient pas fixées par un décret, ainsi qu'en a décidé la commission spéciale, les recommandations d'âge ne pourraient être que très générales et les praticiens de l'assistance médicale à la procréation, auxquels il reviendra concrètement d'apprécier si les personnes qui les consultent « remplissent des critères d'âge », seront mis en difficulté. Il appartient certes au législateur de fixer les règles et d'encadrer la pratique dont nous débattons, mais il convient également

Le Gouvernement ne souhaite pas ouvrir la porte à de telles dérives et revient, par cet amendement, à un cadre rigoureux qui sera validé par les professionnels concernés puisque le décret sera pris après avis de l'Agence de la biomédecine qui les consultera.

Pour faire un peu de philosophie, cela rappelle Karl Popper : il y a une règle du jeu, mais il doit y avoir du jeu dans la règle. Le dispositif que nous proposons garantit ce jeu dans la règle dans de bonnes conditions. La parole est à M. le secrétaire

amendement. Vous souhaitez qu'il soit proposé aux femmes de réaliser une autoconservation d'ovocytes dans le même temps que le prélèvement d'ovocytes en cours de fécondation. Nous pouvons comprendre votre démarche au bénéfice des femmes qui s'engagent dans ces parcours longs et difficiles. De fait, celles qui présentent une insuffisance ovarienne débutante souhaitent parfois faire une préservation de fertilité avant ou pendant la conservation pour augmenter les chances d'avoir plusieurs enfants. Par ailleurs, ainsi que vous l'évoquez, si une femme a conservé des ovocytes, elle pourra les utiliser ultérieurement en formant un nouveau couple avec un autre homme ; de plus, ces ovocytes seront de meilleure qualité puisque prélevés alors qu'elle était plus jeune. Pour autant, cette pratique peut, selon nous, induire une perte de chances pour la femme, tant de la fécondation que de l'autoconservation. Cette dernière, en effet, ne portera que sur peu d'ovocytes et ne garantira donc pas un stock suffisant pour préserver correctement la fertilité. Si cette perte de chances est de plus en plus limitée grâce à l'amélioration des techniques et à la vitrification ovocytaire, notamment, elle reste cependant

la ponction ayant bénéficié au process d'autoconservation évitera, du coup, que le corps de la femme soit à nouveau sollicité en cas d'échec de cette implantation. Nous sommes